Nous le savons tous, l'illectronisme est étroitement lié à la fracture numérique. Celle-ci s'observe particulièrement dans l'inégale couverture numérique dont souffrent spécifiquement les territoires ruraux et les outre-mer. Je prends un exemple concret, la Guyane : ce département ultramarin abrite un centre de recherche spatiale et une base de lancement française

fins d'évaluer l'exclusion numérique et les usages de leurs compétences numériques par les citoyens. Il enjoint le Gouvernement à définir un « référentiel commun d'évaluation des capacités numériques » par décret pris en Conseil d'État. Or le cadre de référence des compétences numériques constitue déjà le référentiel commun desdites compétences, de sorte qu'il serait surabondant d'en élaborer un second.

ces compétences sont déjà évaluées par l'éducation nationale en fin de collège et au lycée par le groupement d'intérêt public Pix. En outre, le programme de la JDC a régulièrement été modifié et densifié au détriment de sa cohérence et de sa réceptivité par un public d'âge compris entre 18 ans et 25 ans. Ajouter un test de compétences numériques viendrait alourdir un programme déjà chargé, sauf à supprimer certains éléments, comme ce fut le cas pour la formation aux gestes de premier secours.

Cela se révèle encore plus pénalisant pour une partie de nos concitoyens qui ne se trouvent pas en mesure d'utiliser internet. Nous devons être guidés par un seul impératif l'amélioration du service rendu aux usagers, au moins le temps nécessaire pour que la transformation numérique des personnes publiques soit totalement assimilée. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet amendement de suppression.

des services publics de choisir les modalités de correspondance avec l'administration, ainsi que les modalités de paiement des services dématérialisés qu'ils souhaitent utiliser. La commission des lois doute que l'inscription de principes généraux symboliques dans la loi apporte de véritables garanties à l'usager. Là aussi, les avancées en faveur de celui-ci passent d'abord par une succession d'actions concrètes adaptées à chaque procédure. En outre, la plupart des administrations proposent déjà plusieurs modalités de paiement et de correspondance au choix des usagers. Ainsi, pour déclarer ses revenus à l'administration fiscale, un usager peut utiliser la voie dématérialisée ou indiquer

explication de vote. La commission des lois et M. le secrétaire d'État doutent que l'inscription de principes généraux symboliques dans la loi apporte de véritables garanties à l'usager. Pourtant, nos grandes lois sont truffées de principes généraux

Or, dans de nombreuses situations, un usager peu à l'aise avec l'outil informatique, mais invité à effectuer ses démarches en ligne, peut en toute bonne foi commettre des erreurs répétées. Il convient donc de prendre en compte cette situation dans une société toujours plus numérisée et hyperconnectée, pour ne pas donner le sentiment que ces personnes en difficulté seraient des usagers de seconde zone. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement la commission sur l'amendement n° 29 ? Cet amendement tend à supprimer la condition selon laquelle le droit à l'erreur prévu par le code des relations entre le public et l'administration ne s'applique que si l'erreur est commise pour la première fois. Néanmoins, cette modification

Son objectif est parfaitement louable, comme celui de tous les autres amendements, à l'heure où les contenus en ligne prennent une place significative. Je pense néanmoins qu'il serait difficile de mettre en place

du numérique, le programme Tech.gouv a pour objectif de permettre à l'État d'accélérer sa transformation numérique. Il doit rendre l'action publique plus proche, plus efficace, plus simple et plus juste pour tous les Français, dans tous les territoires. La feuille de route « Numérique et environnement » rehausse cette ambition, en proposant une stratégie de maîtrise de l'impact environnemental du numérique et de ses effets. Elle invoque l'exigence d'exemplarité de l'État pour la mise en oeuvre d'un numérique responsable à l'échelle du territoire. Dans le cadre du plan de relance, il est prévu de poursuivre et d'amplifier ces actions, qui concernent l'ensemble des administrations. L'écoconception des services numériques vise à maximiser l'impact positif du numérique sur notre société ; elle doit contribuer à une meilleure maîtrise de l'empreinte environnementale des secteurs numérisés. C'est pourquoi j'ai déposé cet amendement qui vise à traduire dans la loi, à travers une exigence d'écoconception des services numériques, la nécessaire articulation entre les principes destinés à garantir une égalité d'accès aux services publics et les engagements environnementaux pour un numérique plus durable. La stratégie nationale bas-carbone doit s'appliquer partout et tout le temps ; sinon, nous n'avancerons pas et nous ne parviendrons pas à baisser nos émissions de gaz à effet de serre.

Plus de la moitié de ces émissions sont dues aux infrastructures de réseaux, notamment aux. La maîtrise de ces émissions n'est donc pas un détail ; c'est même une marge de manoeuvre significative pour réduire le total de notre empreinte environnementale à l'échelle nationale. Cette empreinte pose également une question de souveraineté nationale.

Ce transit par des serveurs étrangers sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise, comme en témoignent les difficultés rencontrées par l'enseignement à distance au début de ce troisième confinement, a un impact fort non seulement sur l'environnement, mais aussi sur notre capacité à maîtriser le trafic de nos données. Puisque l'article 6 traite des sites internet publics et donc de données potentiellement confidentielles et sensibles relatives aux citoyens, cette maîtrise y est d'autant plus nécessaire. L'impact environnemental n'est pas une lubie des écologistes, puisque le Gouvernement lui-même intègre pleinement cette nécessité de maîtriser cet impact environnemental dans la mise en oeuvre d'un numérique responsable à l'échelle du territoire En témoigne la feuille de route « Numérique et environnement » de l'État et, plus largement, la stratégie GreenTech pour toutes les administrations. Mes chers collègues, inclusivité et respect de l'environnement vont de pair.

dans ce texte ; les modalités de ce référentiel seraient précisées par décret. Le numérique est un fer de lance de la transition écologique ; c'est bien vers quoi cet amendement tend.

de leurs auteurs, à savoir réduire l'empreinte environnementale des sites internet et des applications utilisées par les administrations. Toutefois, l'utilisation du seul terme « écoconception » n'est pas suffisante pour fixer de véritables objectifs

et non aux autres administrations, notamment celles des collectivités territoriales. À ce titre, l'amendement tend à supprimer les dispositions pénales prévues par cet article, puisque le montant des pénalités aurait été reversé au budget général de l'État. Enfin, je vous y propose la suppression de la référence aux modalités de saisine alternative. Le principe de saisine alternative semble en voie d'être satisfait par le développement des maisons France Services et la généralisation, dans la plupart des procédures, d'une voie de contact téléphonique.

la ministre de la transformation et de la fonction publiques publie tous les trimestres un observatoire de la qualité des démarches en ligne. Dans cet outil, ces 250 démarches sont évaluées selon plusieurs critères de qualité,

Associer des personnes en situation de handicap à la conception des sites, ainsi que dans les phases de tests et tout au long de la vie du site, permettrait d'éviter ces situations de discrimination.

dans le cadre du plan de relance, Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques a annoncé qu'une enveloppe de 32 millions d'euros serait dédiée à l'amélioration de l'accessibilité et de l'ergonomie des démarches, avec des résultats très concrets.

ce même article 7, puisqu'il sanctionne les manquements aux règles relatives à l'accessibilité numérique et non plus seulement l'absence de mention visible sur la page d'accueil précisant si le site internet est conforme ou non à ces règles. Quel

Cet amendement tend à supprimer l'article 8, qui crée un chèque-équipement numérique afin d'équiper les ménages démunis en terminaux numériques et un fonds de lutte contre l'exclusion numérique, géré par l'Agence nationale de la cohésion des territoires Le Gouvernement prend d'ores et déjà en compte la problématique de l'exclusion numérique dans le cadre de sa stratégie de dématérialisation des services publics et de son plan de relance à travers lequel il y consacre 250 millions d'euros. Les deux aides prévues à l'article 8 risquent de n'être que des coquilles vides en l'absence de garanties de financement et d'articulation avec les dispositifs existants. Par ailleurs, la centralisation des crédits relevant de la lutte contre l'exclusion numérique dans un fonds géré uniquement par l'Agence nationale de la cohésion des territoires pourrait nuire aux nombreuses initiatives locales et nationales, qu'il s'agisse d'aides financières ou d'infrastructures qui prennent déjà en compte les spécificités territoriales.

l'article 9, qui prévoit les modalités de financement du fonds de lutte contre l'exclusion numérique créé à l'article 8. Ces dispositions ne peuvent relever que d'une loi de finances, conformément aux articles 34 de la Constitution et 34 de la loi

ne relèvent pas du domaine de la loi. Elles nécessiteraient simplement que soient complétées les dispositions réglementaires actuellement applicables.

bénéfice de ceux qui, pour des raisons géographiques ou financières, en sont aujourd'hui privés. Ces solutions offrent des opportunités qu'il serait intéressant d'étudier afin d'en connaître la portée. nous demandons que soit remis au Parlement un rapport sur les bénéfices sociaux et les conséquences environnementales des services d'accès gratuit à internet haut débit proposés par les collectivités territoriales, ainsi que sur l'opportunité de leur généralisation.

qui prévoit que soit désigné, au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un « référent en charge de l'inclusion numérique ». Une telle création peut être opportune en fonction des situations locales, mais il n'est pas pertinent d'en faire une obligation juridique pour chaque EPCI. Il convient de laisser les collectivités territoriales et leurs groupements s'adapter à leurs besoins propres.

dématérialisées à la place des usagers. Plus la dématérialisation s'accélère, plus la demande d'assistance numérique croît. Or, selon ce même rapport d'information sénatorial, moins de 10 % des intervenants sociaux ont reçu une véritable formation au numérique. Il apparaît donc cohérent avec une politique réelle de lutte contre l'exclusion numérique de prévoir que les instituts régionaux du travail social délivrent une formation obligatoire à la médiation numérique pour permettre aux travailleurs sociaux d'accompagner au mieux les publics, ainsi que pour pouvoir orienter les personnes en difficulté face au numérique vers des offres de formation existantes. ? Cet amendement tend à former les travailleurs sociaux à la médiation numérique afin qu'ils viennent en aide aux personnes en difficulté dont ils ont la charge. Si je partage l'objectif de l'amendement qui tend à venir en aide aux personnes en difficulté face au numérique, il semble toutefois difficile de mettre en oeuvre une telle mesure sans concertation avec les représentants de ce secteur.

Cet amendement vise à supprimer l'article 12, qui prévoit la prise en compte, à côté de l'illettrisme et de l'innumérisme, de l'illectronisme parmi les priorités nationales en matière d'éducation. Cet article est essentiellement symbolique, puisqu'il ne prévoit ni obligation claire ni objectif tangible. La prise en compte de l'illectronisme aurait donc une portée normative limitée. Elle le serait d'autant plus qu'il n'existe pas de définition claire de ce néologisme.

La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle. Dans ce cadre, cette collectivité contribue notamment à la lutte contre l'illettrisme sur le territoire de la région, en organisant des actions de prévention et d'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences. Cet amendement vise à ajouter la lutte contre l'illectronisme à celle contre l'illettrisme. Quel

au même titre que l'illettrisme. Il ne s'agit pas d'un cavalier, mais les travaux que j'ai conduits ne me permettent pas de juger du bien-fondé de cet ajout. La connaissance des outils numériques de base est devenue une clé indispensable pour accéder au marché de l'emploi.

Cet amendement tend à supprimer le 1° de l'article 13, qui modifie le contenu des enseignements dispensés par les instituts nationaux supérieurs

il nous a été répondu par le Gouvernement que le choix des logiciels se faisait en fonction de l'appétence des fonctionnaires pour des systèmes très professionnels et très coûteux et que c'était pour cette raison que les logiciels libres

de cette argumentation. C'est pourquoi nous proposons une formation spécifique aux logiciels libres pour tous les fonctionnaires, afin qu'ils orientent de façon intelligente les choix de l'administration, puisque celle-ci semble

pour maintenir la continuité pédagogique pendant les périodes de confinement. Cette crise sanitaire a révélé l'importance de l'accès à des équipements et à une connexion internet tout autant que l'hétérogénéité des compétences numériques des enseignants. environnemental (CESE) préconise que l'État et les collectivités territoriales engagent des politiques publiques de coconstruction dans le domaine du numérique éducatif, s'appuyant sur des orientations nationales claires, ambitieuses et compatibles avec les objectifs de développement durable. Cet amendement vise à introduire dans la formation numérique des enseignants et des étudiants du supérieur une sensibilisation à son empreinte environnementale, afin que ces publics soient en capacité d'appréhender les enjeux du numérique à la fois comme un outil et comme un défi pour la transition carbone et la résilience de notre société.

17 tendent à compléter l'article 13 afin que la formation au numérique délivrée aux étudiants et aux enseignants comprenne une sensibilisation à l'empreinte environnementale du numérique et aux usages responsables. Si le contenu de ces amendements n'est pas purement réglementaire, ils tendent à modifier l'alinéa 2 que nous avons souhaité voir supprimer pour ce motif. Par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements. L'amendement n° 40 vise à préciser que les formations visées par l'article 13

de la mission du service public du numérique éducatif qui a été créé par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, auquel contribue un opérateur qui est le réseau Canopé. Par ailleurs, l'organisation de la formation continue des professeurs est de la responsabilité de leur employeur et du recteur dans chaque académie- les Inspé

Merci

dans le cadre du plan de relance à hauteur de 150 millions d'euros. Au total, six dispositifs de sensibilisation, de formation et d'accompagnement seront mis en oeuvre à court terme

Cette disposition n'est pas opérationnelle, puisqu'elle ne détermine pas le jour d'entrée en vigueur des dispositions du texte. Par ailleurs, cet article serait contradictoire avec l'article 9, qui modifie la stratégie nationale d'orientation de l'action publique annexée à la loi pour un État au service d'une société de confiance (Essoc), qui sera caduque dans huit mois. En conséquence, la commission des lois considère que les dispositions de l'article 15 ne sont pas adaptées et qu'il reviendra au Sénat et à l'Assemblée nationale d'affiner ces dispositions transitoires au cours de la navette parlementaire, en fonction des dispositions adoptées . Quel

au bénéfice des Français de l'étranger. Supprimer le « droit au guichet » et le choix des modalités des saisines de l'administration, alors que nos concitoyens ne cessent de rencontrer des obstacles

Social Européen, la discussion de la proposition de loi visant à moderniser et faciliter la procédure d'expropriation de biens en état d'abandon manifeste,

monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je tiens d'abord à saluer l'action de Jacques Mézard, premier signataire de la proposition de loi, en faveur de l'aménagement du territoire, en particulier des villes moyennes, considérées comme des points d'équilibre stratégiques après une période de métropolisation effrénée. est le sens du programme Action coeur de ville, qui vise à revitaliser les centres des 222 villes moyennes sélectionnées. D'autres programmes sont venus ultérieurement compléter cette démarche. Nos territoires recèlent un potentiel de développement indéniable. Le départ de nombre de nos concitoyens des métropoles vers des villes à taille humaine, à la suite de la crise sanitaire et du recours accru au télétravail, démontre que ces villes n'ont jamais cessé d'attirer en raison du cadre et de la qualité de vie Pour accompagner ce rééquilibrage de l'espace, les collectivités locales doivent s'adapter en créant de l'habitat et en favorisant l'implantation d'activités économiques et de services publics là où ils tendaient à disparaître. En somme, ce rééquilibrage se traduira par l'éveil des communes dont les centres-bourgs sont peut-être dégradés ou qui comprennent des bâtiments et des terrains en mauvais état, pouvant ressembler par endroits à de véritables dépotoirs. L'objectif de la présente proposition de loi est d'accompagner la redynamisation de ces collectivités par la mobilisation des biens immobiliers et des terrains existants, mal optimisés du fait du désintérêt de certains propriétaires, qui, pour des raisons diverses, parfois légitimes, les ont délaissés. L'acquisition du foncier par les collectivités locales a également pour vertu d'être compatible avec la lutte contre l'artificialisation des terres en promouvant une gestion rationnelle du foncier. Celui-ci se faisant rare et cher, nous avons considéré utile de faciliter cette acquisition, en modifiant la procédure d'expropriation des biens en état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Créée par la loi du 2 août 1989 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles, la procédure simplifiée d'expropriation pour état d'abandon manifeste, plus allégée et moins coûteuse qu'une procédure d'expropriation de droit commun,

ou aux conseils départementaux de se substituer à la commune sur demande du maire ou en cas d'inaction de la commune dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste. (ÉLAN) a permis d'engager cette procédure sur les parties d'un immeuble situé dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, lorsque des travaux ont condamné l'accès à cette partie. Cette procédure concerne les immeubles ou parties d'immeuble, les voies privées grevées d'une servitude de passage public, les terrains et installations, sans occupant à titre habituel et non entretenus, situés dans le périmètre d'agglomération de la commune. n'aura pas à établir l'existence d'un risque pour la sécurité publique. Elle sera uniquement tenue d'indiquer la nature des désordres affectant le bien. D'après la jurisprudence, le fait qu'un terrain en friche serve d'entrepôt ne constitue pas une motivation suffisante. cette procédure est simplifiée, elle n'en demeure pas moins entourée de formalités et d'étapes telles que : la recherche active des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ; une large information du propriétaire et du public dans des délais suffisants ; l'établissement d'un procès-verbal provisoire et d'un procès-verbal définitif la constitution d'un dossier d'expropriation simplifié contenant une évaluation sommaire des coûts, une identification précise du bien et le plan parcellaire des terrains et des bâtiments ; la validation du projet par le préfet ; la transmission du dossier au juge de l'expropriation. Cette procédure est également entourée de garde-fous : elle ne peut s'appliquer qu'aux biens situés dans le périmètre d'une agglomération et au profit de certaines personnes et d'organismes publics et elle doit avoir pour seule finalité soit une opération liée à l'habitat, soit une opération d'intérêt collectif relevant de la restauration, de l'aménagement ou de la rénovation. La présente proposition de loi vise à apporter des modifications à la marge, en permettant d'exproprier des biens situés en dehors du périmètre d'agglomération, le droit actuel pouvant en effet entraver l'expropriation de corps de fermes situés en bordure des voies publiques. Elle prévoit également d'étendre les finalités de son utilisation en vue de constituer des réserves foncières. Enfin, elle permet à la commune de désigner l'EPCI comme destinataire du bien plus en amont de la procédure. Mes chers collègues, l'objectif premier de cette procédure n'est pas tant l'expropriation que la cessation de l'état d'abandon manifeste du bien. Il est avant tout de mettre fin à des situations de blocage qui s'enlisent. Les propriétaires sont tout d'abord invités à sortir de l'inertie. Ils disposent de trois mois à compter de l'établissement du procès-verbal provisoire pour réagir. Ils peuvent s'engager à réaliser des travaux dans un délai fixé par une convention conclue avec la commune. L'atteinte au droit de propriété est donc limitée et proportionnée grâce à une procédure qui n'est pas dénuée de risques juridiques, si elle n'est pas scrupuleusement respectée. Le droit de propriété est garanti pour la bonne raison qu'il ne peut y avoir d'expropriation que pour cause d'utilité publique. Comme dans le droit commun, le projet ne pourra être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente. Le juge continuera pour sa part d'appliquer la théorie du bilan, en mettant en balance les coûts et les avantages de l'opération, comme il a coutume de le faire depuis l'arrêt du Conseil d'État du 28 mai 1971. Prenant en compte les spécificités locales, nous avons estimé que la priorisation sur les opérations liées au logement, prévue dans le texte initial, ne devait pas être imposée de manière uniforme. C'est la raison pour laquelle nous avons suggéré au rapporteur de préserver l'application de la procédure simplifiée d'expropriation à l'ensemble des opérations d'intérêt collectif qui en bénéficient actuellement. Cette priorisation ne pouvait avoir de sens dans les communes qui ne connaissent pas de difficultés en matière de logement, celles qui sont en situation de déprime démographique et pour lesquelles la création d'équipements collectifs ou la valorisation économique des biens, reconnue par la jurisprudence, aurait davantage d'intérêt. Je remercie donc le rapporteur d'avoir modifié le texte en ce sens. Nous regrettons cependant que l'amendement que j'avais déposé visant à rétablir la possibilité

attendue par les élus locaux qui s'engagent dans une politique volontariste d'aménagement de leur territoire afin de recréer des bassins de vie. Le groupe du RDSE vous invite à soutenir cette démarche afin de compléter les outils juridiques dont disposent les maires pour concrétiser leurs projets d'intérêt local.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi visant à moderniser et faciliter la procédure d'expropriation de biens en état manifeste, déposée par notre ancien collègue Jacques Mézard- je le salue -, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, et inscrite à l'ordre du jour de l'espace réservé au groupe du RDSE. Cette proposition

Comme vous le savez, il s'agit de l'une des procédures exorbitantes permettant aux communes d'accéder à la propriété en dehors de toute cession à titre onéreux, au même titre que les dons et ou l'acquisition des biens sans maître. La procédure de reconnaissance d'état d'abandon manifeste est originale, puisque le transfert de propriété au bénéfice de la commune n'est pas sa seule finalité. Dans un premier temps, ce transfert est un moyen de pression sur le propriétaire, qui est invité à mettre fin à l'abandon manifeste de son fonds une fois que celui-ci est constaté par le maire. Ce transfert de propriété n'intervient que dans un second temps, si le propriétaire ne s'exécute pas. En ce sens, il peut s'agir pour le maire d'une alternative intéressante aux mesures de police administrative spéciale en matière d'habitat insalubre ou d'immeuble menaçant ruine, s'il souhaite que la commune s'approprie le bien. Je remercie donc le groupe du RDSE d'avoir déposé ce texte, car cette procédure répond véritablement à une problématique souvent rencontrée par les maires, qui doivent se substituer aux propriétaires défaillants pour effectuer des travaux sans pour autant parvenir à obtenir un quelconque remboursement de leur part. Elle peut donc être perçue comme une alternative aux astreintes administratives prévues par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique afin d'inciter le propriétaire à mettre lui-même en oeuvre les travaux imposés par des mesures de police administrative spéciale.

La première tendait à supprimer la condition selon laquelle la parcelle concernée doit se situer à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. La procédure pourrait donc concerner des biens sur l'ensemble de son territoire. La deuxième visait à permettre à la commune de prévoir, dès le stade du procès-verbal définitif, que l'expropriation se fasse au profit d'un EPCI, sans attendre le stade de la constitution du dossier. Enfin, la dernière tendait à ouvrir les catégories de projets pouvant donner lieu à déclaration d'état d'abandon manifeste par le conseil municipal, mais à restreindre ensuite ceux de ces projets qui pourraient donner lieu à expropriation simplifiée. Seuls les projets en lien avec l'habitat auraient alors pu ouvrir droit à expropriation simplifiée avec, le cas échéant, la possibilité de constituer une réserve foncière en ce sens. La commission des lois a largement souscrit à la volonté des auteurs de la proposition de loi de simplifier cette procédure pour en améliorer l'efficacité. Ce souhait est d'ailleurs partagé par le Gouvernement, puisque l'article 18 de l'avant-projet de loi dit 4D contient précisément des mesures allant en ce sens. La commission des lois s'est également montrée très favorable à la suppression de l'exigence relative au périmètre d'agglomération de la commune, car cela facilitera évidemment l'accès des communes au foncier de leur territoire.

Je pense qu'il s'agit d'une véritable opportunité qu'il nous faut saisir. Enfin, la commission a été très favorable à ce que la commune puisse faire bénéficier l'EPCI de l'immeuble exproprié dès le début de la procédure, sans remettre en cause la possibilité qui lui est laissée de reprendre une procédure engagée par une commune, mais non conduite à son terme. En revanche, en accord avec le groupe du RDSE, la commission des lois n'a pas été favorable à la modification technique qui tendait à ouvrir les catégories de projets pouvant donner lieu à déclaration d'état d'abandon manifeste, mais à restreindre ensuite ceux de ces projets qui auraient pu donner lieu à expropriation simplifiée. simplifiée. La modification proposée dans la proposition de loi initiale n'allait pas dans le sens présenté dans l'exposé des motifs, puisqu'elle limitait les cas permettant une expropriation simplifiée aux seuls projets en lien avec l'habitat. l'habitat. La jurisprudence nous a montré qu'en l'état actuel du droit un conseil municipal peut déclarer une parcelle en état d'abandon manifeste pour construire, par exemple, un chantier naval, en passant par une expropriation simplifiée, puisqu'il s'agit d'un projet d'intérêt collectif. Avec la proposition de loi initiale,

Les élus locaux ne ménagent pas leurs efforts pour que leurs villes et leurs centres-bourgs soient attractifs. La qualité du cadre de vie est un facteur essentiel de succès et d'attractivité. Cet engagement est, au fond, l'une des premières marques d'attachement à notre patrimoine et à ses habitants. Or chacun d'entre nous a en tête, dans son coeur de ville et de village, un bien abandonné- souvent plusieurs, d'ailleurs -qui se dégrade. Ce sont des verrues- il n'y a pas d'autres mots -, qui peuvent parfois mettre en péril tous nos efforts pour rénover un centre-ville. Je tiens à préciser que ces phénomènes ne se situent pas que dans les centralités. L'entretien de ces biens et, le cas échéant, leur récupération pour conduire les opérations de réaménagement constituent souvent un facteur clé d'une stratégie de redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. Le dispositif relatif aux biens en état d'abandon manifeste du code de l'urbanisme le permet, bien souvent avec succès. Pour autant, le nombre important de biens qui semblent abandonnés doit nous interpeller sur ce dispositif pour l'améliorer. Il s'agit d'un sujet d'actualité, alors que l'Assemblée nationale examine en ce moment même le titre IV du projet de loi dit climat et résilience, dédié à l'artificialisation des sols. En effet, nous devons freiner l'étalement urbain, dont nous mesurons chaque jour les conséquences non seulement écologiques, avec la disparition des terres, lesquelles stockent tout de même 10 % de nos gaz à effet de serre, et la perte de biodiversité, économiques et sociales du fait de l'éloignement de l'habitat des lieux d'activités et de services et de l'autosolisme contraint, de plus en plus coûteux pour beaucoup de nos concitoyens, généralement les plus modestes. Ce phénomène n'est pas pour rien dans la dévitalisation de nos centres-villes et centres-bourgs. Nous ne pouvons y parvenir qu'en modifiant durablement la manière dont nous aménageons le territoire, ce qui nécessite d'intervenir sur deux sujets essentiels. Recycler les zones déjà urbanisées doit devenir plus facile que de faire de l'étalement urbain. C'est l'un des objets de cette proposition de loi qui vise à faciliter la récupération des biens en état d'abandon manifeste. Il nous faut aussi rendre nos zones urbaines désirables, agréables à vivre. C'est indispensable, car habiter en périphérie des villes- à proximité, mais pas trop près quand même -, est une préférence partagée par la majorité des Français.

Le Gouvernement est mobilisé depuis quatre ans dans l'objectif de revitaliser nos territoires, nos petites villes et nos villes moyennes. Il s'agissait d'ailleurs de l'un des principaux engagements de Jacques Mézard, qui avait donné le coup d'envoi avec Action coeur de ville : 222 villes, 5 milliards d'euros et de nombreux outils pour redynamiser et rénover en profondeur nos centres-villes. Les résultats sont là

En parallèle, nous accompagnons la redynamisation économique grâce au programme Territoires d'industrie et aux sites clés en main pour faciliter la réinstallation d'entreprises sur des friches urbaines. Nous accompagnons également la transition numérique grâce au plan France Très haut débit, qui permettra de couvrir l'ensemble du territoire dès l'année prochaine. Enfin, nous remettons des services publics, grâce à France Services. Il nous faut en effet mobiliser tous les leviers pour que la redynamisation des territoires, qui profite en ce moment d'une dynamique favorable du fait de la crise sanitaire, soit véritablement une tendance de long terme. Le projet de loi dit 4D, qui sera présenté ici même au mois de juillet prochain, entend poursuivre cet effort. Nous allons notamment favoriser l'accès au dispositif clé pour l'attractivité des territoires : l'opération de revitalisation des territoires (ORT). Nous avons également prévu de traiter la question des biens abandonnés en réformant la procédure des biens sans maître

cette procédure doit pouvoir être mobilisée pour constituer des réserves foncières- c'est un préalable pour conduire les opérations de réaménagement de nos centres-villes et centres-bourgs. Elle doit aussi pouvoir s'appliquer sur l'ensemble de la commune- si de nombreux biens sont en centre-ville, il en existe aussi en périphérie. Tous les biens « récupérables » doivent pouvoir faire

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la mobilisation du foncier constitue un enjeu majeur pour les maires, en particulier dans le tissu rural, afin de favoriser le développement de leur commune et l'implantation d'activités économiques et de services publics, mais aussi de répondre à la demande croissante de logements. L'objectif de cette proposition de loi est d'accompagner et de soutenir la revitalisation des communes face au problème croissant de la sous-optimisation des biens immobiliers et des terrains abandonnés par leurs propriétaires. La procédure d'expropriation des biens en état d'abandon manifeste, exposée au sein du code général des collectivités territoriales, permet à la commune, à l'intercommunalité ou au conseil départemental de se saisir, sous réserve de l'inaction du propriétaire trois mois après après sa mise en demeure, des biens qui ne sont manifestement plus entretenus. Cette procédure simplifiée peut être réalisée sans enquête publique. Cette proposition de loi vise à corriger des dysfonctionnements dans la mise en oeuvre de cette procédure, tout en ne portant qu'une atteinte limitée au droit de la propriété, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle, et ce dans le respect du cadre juridique existant grâce aux diverses garanties procédurales prévues et au contrôle du juge en bout de chaîne.

Elle permettra également d'améliorer l'esthétique des paysages, dont les maires se font les garants. L'actuelle limitation ne se justifie pas : un bien abandonné reste un bien gênant, où qu'il se trouve. Cette situation Cette situation reste préjudiciable, notamment lorsque les parcelles se situent à l'entrée des communes. Au-delà de la valorisation du territoire, la proposition de loi concourt également à aider les maires soumis à à l'objectif de zéro artificialisation des sols dans le cadre de la transition écologique que notre société doit opérer. De même, elle participe à un effort de simplification partagé par le Gouvernement et va dans le sens de l'article 18 de l'avant-projet de loi dit 4D qui devrait, je l'espère, être examiné prochainement par le Parlement. Enfin, je profite de cette tribune pour évoquer la procédure d'acquisition d'un bien sans maître qui reste excessivement longue et qu'il serait également pertinent de dépoussiérer. En effet, lorsqu'il est connu, le décès du propriétaire sans héritier doit être constaté depuis plus de trente ans. Si le propriétaire n'est pas connu, il demeure possible de récupérer le bien, lorsque les taxes foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de trente

qui s'engagent dans une action volontariste de redynamisation de leurs territoires.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens à saluer le texte qui nous rassemble ce soir. Il s'agit d'une initiative parlementaire bienvenue de nos collègues du qui vient concrètement soutenir nos maires dans leurs opérations d'aménagement en simplifiant un outil pertinent pour obtenir le foncier nécessaire à la réalisation de leurs opérations d'aménagement. Loin de se résoudre à laisser nos villes, mais surtout nos villages, en décrépitude, les auteurs de cette proposition de loi accompagnent un mouvement de fond, et un urbanisme rénové (ALUR) de 2014, visant à permettre un renouvellement de la ville sur elle-même. Nous savons que l'urbanisme et l'aménagement sont les deux versants de la vitalité d'un territoire. C'est justement par cet urbanisme et par cet aménagement que nous pourrons optimiser l'occupation d'un territoire et renforcer son dynamisme, particulièrement au centre des agglomérations, dans le strict respect du droit de propriété.

En supprimant la condition selon laquelle le fonds concerné doit se situer à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune, ce texte prend en compte la réalité de la diversité de nos communes- parcelles isolées

qui ne souhaite pas restreindre l'accès à la procédure d'expropriation simplifiée afin de donner plus d'ampleur à cette procédure bienvenue et de permettre au plus grand nombre d'élus locaux de se l'approprier. Cette initiative parlementaire de qualité anticipe, à elle seule, deux discussions que nous aurons dans les prochains mois dans cet hémicycle sera relative au projet de loi dit 4D, puisque l'article 18 de son avant-projet rejoint le premier thème de l'article unique de la présente proposition de loi en élargissant la procédure d'acquisition des biens en état d'abandon manifeste

ou en densifiant le tissu déjà urbanisé. Alors que l'artificialisation des sols a augmenté de 70 % quand la population croissait de 20 %, la présente proposition de loi est un point de départ bienvenu de ce débat.

En effet, il y a là un vrai enjeu pour de nombreuses communes, en particulier dans nos territoires ruraux et périurbains. Aussi, je tiens à saluer l'initiative du groupe du RDSE, qui nous donne l'occasion d'en débattre et de légiférer ce soir. Cette proposition de loi vise à lutter contre les situations d'abandon de biens immobiliers auxquelles nos élus locaux sont confrontés dans leur commune. Nous avons toutes et tous, dans nos circonscriptions, des exemples pour illustrer cette réalité friches, hangars, bâtisses à l'abandon ... Autant de verrues disgracieuses qui nuisent à nos paysages. Face à cette triste réalité, nos collègues maires rencontrent de grandes difficultés, les outils juridiques existants s'avérant souvent insuffisants. Cette proposition de loi vise donc à compléter et à parfaire notre arsenal juridique. À côté des outils permettant de lutter contre l'habitat insalubre et les immeubles en ruine ou en situation de péril, il s'agit de doter nos élus locaux d'un nouveau levier pour contraindre un propriétaire à remédier à l'état d'abandon de son immeuble ou, à défaut, de procéder à l'expropriation en simplifiant la procédure. Aujourd'hui, la dépossession au profit des communes est doublement limitée. La première restriction est géographique : les biens dont une commune peut demander l'expropriation doivent se situer dans le périmètre dit d'agglomération. La seconde concerne l'objet des situations pouvant légitimer une expropriation. Ces restrictions entravent, hélas !, l'action des élus locaux. C'est à ce besoin de liberté, de souplesse et d'efficacité dans l'action locale que veut contribuer cette proposition de loi. Dans un premier temps, les auteurs de ce texte se sont attaqués à la restriction géographique des procédures simplifiées d'expropriation. Cette limitation avait été votée dans la loi de 1989, comme cela a été rappelé, afin que ce dispositif ne puisse être employé pour des terrains laissés provisoirement en friche dans des zones agricoles. agricoles. Cette restriction se justifiait juridiquement dans la mesure où ces parcelles auraient pu faire l'objet d'une procédure d'expropriation. Dans les faits, ce risque est extrêmement limité. Cette méfiance, voire cette défiance, à l'égard des maires ne se justifie objectivement pas. Les auteurs de ce texte proposent donc de supprimer cette restriction géographique pour les biens se trouvant en dehors du périmètre d'agglomération de la commune. Une telle modification du droit devrait permettre aux maires de se saisir de biens susceptibles de générer des difficultés, à l'image de certains corps de ferme situés en bordure des voies publiques. Faire sauter ce verrou géographique est souhaitable, il est donc bienvenu. Cette première disposition relève du bon sens et recueille le soutien du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Dans un second temps, les rédacteurs de cette proposition de loi ont souhaité élargir la liste des destinations des biens faisant l'objet d'expropriation en raison de leur état d'abandon manifeste. Le droit positif prévoit que l'expropriation doit avoir pour objet soit la construction ou la réhabilitation à des fins d'habitat soit un intérêt collectif relevant d'une opération de restructuration, de rénovation ou d'aménagement. L'inscription de ces motifs dans la loi restreint les possibilités des élus locaux d'user de la procédure simplifiée d'expropriation pour des projets tournés vers la valorisation économique de leur territoire.

Ce choix rédactionnel nous avait interpellés en ce qu'il fragilisait juridiquement le texte. En effet, si aucun motif n'était inscrit dans la loi, l'expropriation aurait pu devenir générale et s'appliquer dans n'importe quelle situation. Elle n'aurait donc plus été réservée aux cas justifiés par l'intérêt général.

de mention expresse de la destination du bien faisant l'objet d'une déclaration d'abandon manifeste aurait donc pu fragiliser le texte. Dans sa grande sagesse, la commission des lois a adopté une rédaction alternative, proposant de compléter la liste des motifs justifiant la constitution d'une déclaration d'abandon manifeste. Notre groupe salue cette initiative qui apporte des garanties juridiques plus solides. La proposition de loi prévoit ensuite qu'une expropriation qui se fait traditionnellement au bénéfice de la commune puisse également se faire au profit d'une intercommunalité. Cette évolution nous semble bienvenue, puisque l'intercommunalité dispose de moyens administratifs, juridiques et financiers plus importants qu'une commune. Il semble donc plus aisé d'enclencher une telle procédure à cette échelle. Vous l'aurez compris, nous partageons la philosophie générale du texte proposé par nos collègues du groupe du RDSE. Les contributions et corrections apportées par la commission des lois ont été de nature à améliorer sensiblement cette proposition de loi. Je salue le rapporteur pour son travail. travail. Les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain sont favorables à l'adoption de ce texte. La parole

Aussi, nous nous félicitons de l'initiative de nos collègues du groupe du RDSE qui vise à faciliter et moderniser la procédure d'expropriation de biens en état d'abandon manifeste. procédure permet aujourd'hui à la commune, à la communauté de communes ou au conseil départemental de se saisir de biens qui ne sont manifestement plus entretenus. Cette procédure simplifiée peut être réalisée sans enquête publique. Ainsi, les expropriations peuvent-elles être réalisées en vue soit de construire des logements sociaux soit de réaliser tout projet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. Cette procédure a été créée pour aider les communes dans leurs efforts de rénovation et de réhabilitation du patrimoine local. Elle permet de traiter, dans le périmètre des agglomérations, les immeubles bâtis ou non bâtis à l'abandon ou en ruine et de favoriser leur réaménagement. proposition de loi concourt à remédier à des dysfonctionnements dans la mise en oeuvre de cette procédure, en apportant des corrections et des simplifications. Ce texte propose ainsi d'ouvrir la procédure aux parcelles situées à l'extérieur du périmètre d'agglomération. Cette avancée facilitera l'accès des communes à l'ensemble du foncier de leur territoire. loi tend à supprimer la limitation des finalités d'utilisation des biens saisis par les collectivités- essentiellement liés à l'habitat aujourd'hui -afin d'offrir davantage de possibilités et de souplesse aux communes. Elle distingue deux régimes pour la mise en oeuvre de la procédure : d'une part, une procédure simplifiée, sans enquête publique préalable, pour les expropriations concernant les biens à l'état d'abandon impliqués dans des opérations en matière d'habitat ou la constitution de réserves foncières en vue de telles opérations d'autre part, une procédure de droit commun, régie par le code de l'expropriation, pour cause d'utilité publique comme la création d'espaces publics, la valorisation d'activités économiques ou la construction d'équipements collectifs. À cet égard, nous approuvons la position de la commission qui a jugé utile de revenir sur la disposition technique qui tendrait à ouvrir les catégories de projets éligibles aux déclarations d'état d'abandon manifeste, mais à restreindre ensuite ceux qui pourraient donner lieu à une expropriation simplifiée. Comme l'a souligné le rapporteur, une telle démarche ferait perdre sa pertinence à cette proposition de loi et les avancées qu'elle permettrait. Par ailleurs, nous sommes d'accord avec la commission qui souhaite ouvrir cette procédure à la constitution de réserves foncières.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme cela a été dit, la procédure d'expropriation des biens en état d'abandon manifeste, prévue au sein du code général des collectivités territoriales, permet à la commune, à l'intercommunalité ou au conseil départemental de se saisir, sous réserve de l'inaction du propriétaire trois mois après mise en demeure, des biens qui ne sont manifestement plus entretenus. La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui cherche à étendre cette possibilité au périmètre global de la commune et à la simplifier, notamment notamment au profit des EPCI. Dans son article unique, le texte prévoit d'élargir la procédure d'expropriation des biens aux parcelles situées à l'extérieur du périmètre d'agglomération,

Le droit limite les finalités d'utilisation des biens saisis par les collectivités soit aux opérations de reconstruction ou de réhabilitation aux fins d'habitat, soit à toute opération d'intérêt collectif relevant de la restauration, de l'aménagement ou de la rénovation. Or la proposition de loi supprime cette limitation, notamment afin de faciliter les projets engagés pour la valorisation économique des territoires, en l'assortissant d'une procédure de droit commun régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans tous ses cas de figure, comme la création d'espaces publics, la valorisation d'activités économiques ou la construction d'équipements collectifs.

une destination agricole ? La procédure actuelle prend tout son sens au niveau de l'habitat. Mais demain, ne pourrions-nous pas craindre qu'une municipalité décide de procéder à l'expropriation d'une friche agricole au pourtour de son agglomération, peut-être pour y construire légitimement des logements, mais peut-être aussi pour y implanter des entrepôts ? L'arrêt de l'artificialisation des sols, voire la désartificialisation, est un levier majeur de la lutte contre le réchauffement climatique. Il peut apparaître mal venu de multiplier les opportunités de faire reculer les zones agricoles. Mes chers collègues, permettez-moi une réflexion. Vous défendez habituellement si ardemment, dans cet hémicycle, le droit de propriété, que nous devrions rester tout aussi prudents dans cette possibilité d'y déroger. d'autant plus que l'acte du procès-verbal d'abandon provisoire est réputé notifié par la publicité locale en mairie et dans les journaux, si la personne en cause ou son adresse n'est pas connue. Je note que ce droit de propriété semble paraître beaucoup plus important à certains, lorsqu'il les incite à s'opposer à la réquisition de biens vides non occupés pour pourvoir à la pénurie de logements que lorsqu'il s'agit de la valorisation d'activités économiques. Le droit français conçoit l'expropriation comme une atteinte exceptionnelle au droit de propriété, mais il semblerait que l'appréciation de l'atteinte exceptionnelle varie selon les situations et les bénéficiaires Le droit de ne rien faire de son bien ne saurait être toléré, quand une collectivité peut y voir une opportunité de développement, mais resterait-il sacro-saint, quand il s'agit de biens construits, finis et entretenus qui pourraient participer à l'hébergement des mal-logés ? ? C'est un vrai problème ! Une autre alerte attise ma prudence. Les possibles dérives, déjà constatées, d'utilisation de la procédure comme un simple levier de développement foncier. La prudence nous impose de voir si un changement de destination à plus ou moins long terme de ces terrains expropriés ne contreviendrait pas à l'esprit de la loi. C'est pourquoi, malgré une compréhension des attentes raisonnables des collectivités sur le sujet, en raison de ces réserves sérieuses face à des risques réels, le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires ne votera pas ce texte.

Elle nous permet d'amorcer un débat sur une procédure qui constitue un levier important pour la valorisation de nos territoires. Je salue à ce titre le groupe du RDSE pour l'inscription de ce texte dans son espace réservé, et plus particulièrement son auteur, Jacques Mézard, qui a siégé, pendant plus de dix années, au sein de cet hémicycle. Il s'agit donc, cela a été dit, de faciliter la procédure d'expropriation des biens déclarés en état d'abandon manifeste. Cette procédure présente un intérêt non négligeable : elle permet aux communes, dans des modalités simplifiées, d'accéder à la propriété et de répondre aux nécessités de leur territoire en matière d'habitat ou d'aménagement. Elle permet dans le même temps de faire cesser des situations dommageables, et parfois ubuesques, dans lesquelles des biens se trouvent vides et dépourvus de tout entretien, sans perspective d'une quelconque évolution de cet état de fait. En souhaitant faciliter l'expropriation des biens en état d'abandon manifeste, la proposition de loi s'inscrit dans la continuité d'autres textes. Je pense notamment à la loi ALUR de 2014 de 2014 et à la loi ÉLAN, adoptée en 2018, qui a rendu automatique le constat d'abandon, dans le périmètre d'une opération de revitalisation, des parties d'immeubles dont l'accès a été condamné par des travaux.

elle introduisait en effet un régime hybride d'expropriation pour les biens en état d'abandon manifeste, présentant le risque d'être plus restrictif et en tout cas source d'incertitudes dans ses effets. En maintenant l'architecture prévue par le code général des collectivités territoriales, la présente proposition de loi s'inscrit en pleine cohérence avec les évolutions successives de la loi. La loi du 23 juin 2011 a en effet créé une procédure spécifique aux biens en état d'abandon manifeste, alors que la législation antérieure leur appliquait le droit commun de l'expropriation pour cause d'utilité publique, plus contraignant et finalement mal adapté aux situations visées. Nous approuvons également les trois apports de la proposition de loi conservés par la commission, qu'il s'agisse de l'extension de la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste au-delà du périmètre d'agglomération de la commune, de l'extension de la procédure simplifiée d'expropriation à la finalité de la constitution d'une réserve foncière et de l'ajout des EPCI comme bénéficiaires potentiels de l'expropriation, dès la phase de déclaration d'état d'abandon manifeste. Cette dernière clarification s'inscrit dans la continuité du droit de suite donné par la loi ALUR aux EPCI. Les deux premières dispositions citées nous paraissent en outre de nature à favoriser les opérations de réaménagement, cela a été dit. Elles sont d'ailleurs inscrites dans l'article 18 de l'avant-projet de loi dite 4D. Les différents textes cités montrent bien que les gouvernements et législateurs successifs se sont intéressés à cette procédure originale, en ce qu'elle permet l'expropriation simplifiée par la collectivité de biens abandonnés, mais qu'elle donne également au maire les moyens, en amont, de contraindre le propriétaire à reprendre en main un bien dégradé et source de nuisances pour sa commune. Cette procédure répond concrètement à une problématique souvent rencontrée par les maires, qui doivent se substituer aux propriétaires défaillants pour effectuer des travaux, sans toujours parvenir à un remboursement. Le groupe RDPI approuve à son tour cette proposition de loi dans l'équilibre qui résulte de son examen en commission. Ce texte ouvre utilement un débat qui devrait se poursuivre lors de l'examen attendu du projet de loi 4D. La parole

répondant à une question orale au Sénat au sujet des procédures d'état d'abandon manifeste et de biens sans maître reconnaissait qu'elles étaient de plus en plus difficiles à mettre en oeuvre et peu utilisées, posant ainsi la question de leur opérationnalité. Cette proposition de loi apporte une évolution positive à la procédure d'expropriation des biens en état d'abandon manifeste. Tout d'abord, je tiens à saluer le travail de simplification accompli par M. le rapporteur François Bonhomme, qui a permis l'adoption de cette proposition de loi à l'unanimité de la commission des lois. Quelle commune ne compte pas, dans l'une de nos régions, de maison vacante ou de terre abandonnée ? Cette situation plus que fréquente suscite désarroi et défaitisme : la propriété privée est sacrée et on ne peut y attenter Pour autant, des moyens existent, qui, sans remettre en cause les fondements du droit de propriété, ouvrent des possibilités pour les communes de remettre en vie un patrimoine en déshérence. Ce mode d'acquisition foncière singulier permet aux maires de faire cesser l'état d'abandon de la parcelle au lieu de multiplier les arrêtés de péril et les dépenses d'entretien jamais recouvrées ; il permet aussi de limiter les risques de squats. Autant de situations qui constituent quelques fois des obstacles à la mise en oeuvre d'une politique d'urbanisme ou peuvent contribuer à la dégradation d'un centre-bourg ancien. Cette proposition de loi constitue donc une avancée par l'élargissement du périmètre d'intervention à tout le territoire de la commune, au-delà de l'agglomération, et lui donne un caractère véritablement opérationnel. Cette simplification est également bienvenue dans le cadre de la crise du logement que nous traversons, avec une baisse alarmante de la construction neuve et l'effondrement du nombre de logements sociaux Si la procédure d'abandon manifeste ne permettra pas de massifier la construction ni de relancer le secteur, il ne faut pas négliger son utilité, puisqu'il est possible, pour une commune, de revendre le bien objet de la procédure à un bailleur social ou à un particulier. L'ajout par la commission des lois de l'objectif de « création de réserves foncières » permettant la réalisation des projets d'aménagement ou d'urbanisme est très encourageant pour les opérations d'urbanisme ou les opérations de revitalisation du territoire, qui nécessitent parfois beaucoup de foncier. La question de la lutte contre l'artificialisation des sols fera débat dans le projet de loi face à ses effets. Aussi, étendre la procédure d'expropriation des biens en état d'abandon manifeste permettra la réappropriation des espaces urbanisés.

Il s'agit de l'identification des héritiers, qui prend du temps et a un coût important pour les communes, tout particulièrement dans les territoires ruraux. Le groupe Les Républicains votera bien évidemment cette proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe du RDSE nous offre de traiter ce soir un véritable sujet communal, un sujet concret, un sujet d'élus, un sujet de petit bourg rural ou de grosse agglomération urbaine. s'agit surtout d'un sujet casse-tête, pour lequel il nous faut des outils réellement opérationnels et efficaces. Nous avons tous, mes chers collègues, rencontré ce type de dossier, celui de la ruine, moche, parfois dangereuse, qui bloque d'autres projets et amène les voisins à venir râler tous les mois dans le bureau du maire. alors un cycle infernal. Il faut se transformer en Sherlock Holmes pour retrouver la piste d'éventuels propriétaires, partis, décédés, divorcés ou expatriés, des fantômes introuvables et désirés, tellement désirés parce qu'ils ont la clé. Parfois, on les trouve, et ils ne font rien, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas : indifférence, procédure en cours, et c'est parti pour des années de casse-tête et de désespoir. L'édifice est une verrue, on finit par ne voir que lui. Depuis peu, alors que les sujets de consommation d'espace prennent de l'ampleur, l'emprise occupée pour rien devient encore plus insupportable. Alors qu'il faut réussir à maintenir le dynamisme démographique sans faire d'étalement urbain, pouvoir « recycler » les biens en état d'abandon manifeste est un vrai enjeu. Mais c'est encore un parcours de l'élu combattant. Pour abréger le suspens, je dirai que le groupe Union Centriste votera pour ce nouvel outil qu'est la proposition Elle intègre à juste titre le fait que les biens en état d'abandon manifeste peuvent se situer en tout point du territoire. Elle lève également les difficultés qui pourraient surgir des partages de compétences entre communes et EPCI. Mais je profite de cette prise de parole pour évoquer les lacunes de la boîte à outils des élus. Si la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, peut désormais être utilisée pour la démolition de bâtiments abandonnés, il faudrait que les services et les élus aient largement connaissance de cette possibilité. largement connaissance de cette possibilité. Pourquoi ne pas la rendre également mobilisable pour les travaux urgents que les municipalités doivent parfois engager en lieu et place des propriétaires défaillants ? ? Dans tous les cas, pour engager les démarches, les maires ou présidents d'EPCI devraient pouvoir bénéficier d'aides financières pour faire face aux divers frais liés aux expertises, aux constats d'abandon, à la publicité et aux autres procédures forcément coûteuses. La finalité de ce texte n'est pas de faciliter l'expropriation, mais de permettre d'envoyer un message musclé aux propriétaires inscrits aux abonnés absents. La finalité est bien de faire disparaître les biens abandonnés Pour ce faire, il faut, vous aurez compris mon message, des lois et des aides financières. Si le groupe du RDSE fait aujourd'hui une gymnastique admirable entre droit de la propriété privée et article 40 de la Constitution, les élus ont vraiment besoin, monsieur le secrétaire d'État, de beaucoup plus.

la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui démontre la volonté du Sénat de simplifier la vie des collectivités territoriales. Nous, sénateurs, sommes en effet régulièrement interpellés par les maires de nos départements sur les difficultés qu'ils rencontrent concernant des immeubles ou des terrains délaissés. À la suite de mes visites dans les communes de Moselle, je peux attester qu'il s'agit d'un sujet récurrent. Il est tout naturel que notre assemblée se soit saisie de cette proposition de loi visant à moderniser et faciliter la procédure d'expropriation de biens en état d'abandon manifeste. La négligence des propriétaires, leur éloignement géographique ou les problèmes successoraux font que ces biens non entretenus se dégradent peu à peu. Face à l'inaction de ces propriétaires, les municipalités se trouvent empêchées d'aménager l'espace pour y accueillir de nouveaux habitants, implanter des services ou valoriser économiquement le territoire.

Engagée par le maire, la procédure permet de déterminer les parcelles, de notifier au propriétaire le procès-verbal établissant l'état d'abandon manifeste et de lui imposer un délai de trois mois pour se manifester. délai, sans réponse ni action de sa part, un procès-verbal permet d'établir l'état d'abandon définitif. Selon une procédure simplifiée, une expropriation peut être engagée, à condition qu'elle ait pour but la construction de logements ou tout objet d'intérêt collectif. La commission des lois et son rapporteur, M. François Bonhomme, ont été favorables à l'esprit général du texte, mais ont souhaité l'améliorer et le conforter. Notre commission a conservé deux points positifs : la levée du « périmètre d'agglomération de la commune qui permettra au maire d'agir sur l'ensemble du territoire, et la possibilité dont disposera l'EPCI de devenir bénéficiaire de l'expropriation. En revanche, afin de clarifier le texte et de le rendre plus cohérent, il n'a pas été jugé utile de retenir les dispositions ayant pour conséquence de ne réserver la procédure d'expropriation simplifiée qu'aux opérations liées à l'habitat. Cela semblait en contradiction avec les objectifs mêmes de la proposition de loi. Le rapporteur a judicieusement élargi la liste des projets permettant la déclaration d'état d'abandon. Il a cependant veillé à ne pas faire bouger les lignes de façon excessive entre la procédure normale, relevant du code de l'expropriation, et la procédure dérogatoire. Il était également important de garantir le respect du droit de propriété, en conservant cette liste au stade de la procédure normale. Je voudrais rendre hommage à l'excellent travail réalisé par le rapporteur de la commission des Lois, M. François Bonhomme. Nous souhaitons que les maires puissent agir plus librement pour aménager l'espace et y accueillir des habitants, des services et des activités économiques, à l'heure où la ruralité connaît une nouvelle attractivité. À cette fin, la proposition de loi, améliorée par les travaux de la commission, constitue un bon véhicule législatif. Elle est aussi un prélude à nos travaux sur le projet de loi 4D, qui sera examiné par le Parlement dans les prochaines semaines. La parole

Tels sont les termes du dix-septième et dernier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pour la première fois, la notion de nécessité publique faisait son apparition dans un texte, qui est désormais de valeur constitutionnelle. Plus de 230 ans plus tard, c'est ce même impératif de nécessité publique qui conduit le législateur à faire évoluer le droit sur le sujet et à renforcer les prérogatives des collectivités en matière d'urbanisme. Les dernières décennies ont été ponctuées d'évolutions majeures et rapides en matière de logement en France, chacune d'entre elles se proposant d'être une réponse aux nouveaux enjeux de transition écologique et de modernisation des territoires : les lois ALUR, puis ÉLAN, la création de l'ANCT, l'Agence nationale de la

Les biens immobiliers laissés à l'abandon, nombreux dans la ruralité comme en ville, sont créateurs d'un certain lot de retombées particulièrement délétères pour les communes. Ces fameux « biens sans maître » immobilisent des parcelles parfois précieuses, là où l'évolution rapide des valeurs foncières recommanderait une valorisation sans délai du terrain. Qu'ils soient localisés à l'entrée ou dans les centres des bourgs, ces biens nuisent à l'attractivité et à l'image globale de la commune. Ils favorisent le développement des squats et des nuisances diverses qui en découlent- insalubrité, vétusté -, sans compter les risques sécuritaires, qui font encore peser sur les épaules des maires une responsabilité périlleuse- danger d'effondrement, non-entretien des installations électriques ou de gaz, etc. À l'heure de la cohésion des territoires et de leur valorisation économique, il s'agit d'une mesure de bon sens que d'enrichir l'arsenal des maires, afin de remédier à ce phénomène. L'élargissement de la compétence d'expropriation à l'ensemble du territoire de la commune, et non plus à son seul périmètre d'agglomération, est une première pierre dans l'édifice de la continuité urbaine des territoires, à plus forte raison à l'heure des fusions de communes et de la montée en compétence des intercommunalités. Assurer le développement du tissu construit entre plusieurs centres-bourgs, le long des axes routiers, sera une façon de se prémunir contre le maintien d'îlots mal connectés et mal urbanisés et d'assurer une plus grande connexion entre les territoires. par M. le rapporteur visant à prévoir le critère de constitution de réserves foncières est un remède judicieux pour pallier la crise du logement et les tensions dans la détermination de nouvelles parcelles constructibles. Enfin, l'inclusion des EPCI dans les bénéficiaires des terrains expropriés est un levier de choix pour soutenir leur montée en compétence. Force est donc de constater la grande plus-value de ces propositions portées par M. Jean-Claude Requier et appuyées par notre collègue rapporteur François Bonhomme.

préciser que la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être prononcée que pour les établissements publics de coopération intercommunale « y ayant vocation », c'est-à-dire ceux qui détiennent une compétence habitat ou aménagement correspondant aux opérations justifiant l'expropriation. D'autre part, il tend à ce que les règles fixant la forme des arrêtés pris par le préfet pour déclarer l'utilité publique de l'immeuble en cause prennent en considération toutes les catégories de bénéficiaires au profit desquels l'expropriation peut être poursuivie.